La séance est reprise. Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

il inclut dans la superficie des parcs de stationnement les voies et cheminements de circulation situés dans le périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties. Or, compte tenu des espaces nécessaires aux manœuvres des poids lourds, dont la longueur peut atteindre 18,35 mètres, il paraît matériellement impossible d’équiper les voies et les cheminements de circulation de ces véhicules en ombrières photovoltaïques. Cette situation est source d’inquiétude pour les professionnels du secteur,

à cette date ; mais la situation d’une conclusion ou d’un renouvellement intervenant entre le 1 juillet 2026 et le 1 juillet 2028 n’est pas envisagée. L’article 26 répare cette lacune, en prévoyant que l’ensemble des contrats dont le renouvellement intervient après le 1 juillet 2026 entrent en vigueur au 1 juillet 2028. La

ainsi que d’un bon de commande au plus tard le 31 décembre 2025. La loi Industrie verte date d’octobre 2023, soit suffisamment tôt par rapport à ces échéances pour permettre aux acteurs concernés d’anticiper le report de l’obligation si tel était leur souhait. était leur souhait. Ainsi, le glissement d’un an pour l’échéance de l’obtention d’un contrat d’engagement et de six mois pour le bon de commande ne nous semble pas nécessaire, dans une perspective concrète d’accélération du développement des installations solaires sur les grands parcs de stationnement.

En effet, la dérogation prévue à l’article 23 de la loi Industrie verte n’a, en pratique, jamais pu être utilisée. Le décret précisant les caractéristiques des panneaux solaires ouvrant droit au report de l’échéance a été publié le 4 décembre 2024, soit moins d’un mois avant le délai limite prévu avant la conclusion d’un contrat d’engagement avec acompte. Le report d’un an de l’échéance est donc nécessaire pour soutenir une filière française de panneaux photovoltaïques

en commission. Le X dispense les collectivités de l’obligation de constituer une régie pour exploiter des installations de production d’énergie renouvelable, au delà de la dérogation déjà existante pour les projets photovoltaïques de moins de 1 mégawatt en autoconsommation. cette disposition entre en contradiction avec le principe selon lequel les usagers n’ont pas à financer les dépenses incombant au contribuable. Le XI uniformise le critère de proximité géographique de l’autoconsommation, étendu à vingt kilomètres pour tous les projets quel que soit le territoire, et supprime le critère de puissance maximale. Le cadre de l’autoconsommation collective étendue est dérogatoire aux principes de fonctionnement du marché de l’électricité. Les conventions d’autoconsommation sont moins protectrices pour les consommateurs que des contrats de fourniture d’électricité classique. Les opérations d’autoconsommation collective étendue induisent des coûts pour le système électrique, qui sont supportés non pas par leurs participants, mais par l’ensemble des utilisateurs du système électrique. Il importe dès lors de limiter la taille de ces opérations, pour garantir une proximité forte entre les différents participants d’une opération d’autoconsommation,

l’article 26 ne supprime pas les critères de puissance maximale et de proximité géographique. Il se contente d’élever au niveau législatif le critère de proximité géographique et de l’uniformiser

ainsi libellé : La parole est à M. Jérémy Bacchi. Le présent amendement vise à lever les incertitudes juridiques freinant le développement des énergies renouvelables, en clarifiant le régime applicable aux panneaux solaires implantés dans des zones naturelles.

Afin de sécuriser ces projets et d’accélérer la transition énergétique, il est proposé de préciser que les zones naturelles accueillant des infrastructures de production d’énergie solaire photovoltaïque, après obtention d’une autorisation de défricher et d’un permis de construire, cessent de relever du régime forestier pour la durée d’exploitation des installations. Monsieur le sénateur, votre amendement vise à exclure du régime forestier les bois et forêts sur lesquels sont implantés les ouvrages nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque. Le régime applicable aux panneaux solaires dans les bois et forêts prévoit que la décision d’autorisation de défrichement comporte des mesures de reconstitution de l’état boisé en fin d’exploitation. Cette obligation

L’implantation de tels ouvrages n’est donc pas incompatible avec le maintien du régime forestier. Le Conseil d’État a ainsi précisé que, dès lors qu’un retour à l’état de forêt est prévu en fin d’exploitation photovoltaïque, le régime forestier doit être maintenu. Sur le fondement de ces éléments, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Ce sous amendement vise à rapprocher la rédaction de l’amendement n° 11 rectifié de celle de l’article 16 de la directive RED III, que l’amendement vise à transposer.

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable avait adopté un amendement prévoyant une telle durée limite en zone d’accélération, dans le cadre de l’examen du projet de loi Industrie verte, sur l’initiative de son rapporteur Fabien Genet. Cette toutefois pas survécu à la navette. Comme pour les amendements précédents, cette durée maximale est prévue par la directive RED III et la France est, là aussi, en retard, puisqu’elle devait transposer cette mesure avant le 1 juillet 2024. Ce délai limite différencié permet également de renforcer les avantages associés à l’implantation des zones d’accélération, dispositif créé par la loi Aper sur l’initiative de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et qui place le

Ces amendements tendent à transposer la directive RED III, en limitant dans la loi les délais d’instruction des projets d’énergie renouvelable. Cette directive prévoit la mise en place de zones d’accélération soumises à une évaluation des plans et programmes, dans lesquelles les projets bénéficieront de procédures d’autorisation simplifiées, avec une exemption d’étude d’impact et des délais réduits. Néanmoins, il est fait référence dans ces amendements aux zones d’accélération définies par l’article L. 141 5 3 du code de l’énergie, issu de la loi Aper, alors que ces deux types de zones sont différents et ne peuvent se substituer l’un à l’autre.

but est d’accélérer les procédures d’autorisation pour la modernisation des installations d’énergie renouvelable. Nous proposons que la procédure d’octroi de l’autorisation n’excède pas six mois pour les projets situés en zone d’accélération et que le délai maximal de l’instruction soit d’un an. soit d’un an. Ce délai pourrait être prolongé de trois mois en cas de circonstances exceptionnelles. L’adoption de cet amendement permettra de respecter les délais fixés par la directive, qui devaient être transposés en législation nationale avant le 1 juillet 2024. Cette mesure répond à une demande urgente de la Commission européenne, qui a insisté sur la nécessité d’adopter ces règles pour faciliter les projets d’énergie renouvelable en accélérant les procédures d’octroi de permis.

Le déploiement de réseaux de chaleur ou de froid renouvelables contribue à la décarbonation et à l’efficacité énergétique, en valorisant les ressources renouvelables, comme la chaleur fatale, la géothermie, la cogénération ou le solaire thermique. Encourager l’analyse du potentiel de valorisation de la chaleur

(EPCI) de plus de 45 000 habitants. Ces collectivités offrent un cadre idéal pour développer et optimiser de tels réseaux, car elles permettent de mutualiser les besoins énergétiques et de diversifier les sources. en effet d’une diversité de besoins énergétiques et de potentiels locaux pour la production énergétique. Cette mesure assurerait une prise en compte efficace des enjeux énergétique par les territoires.

retirerait les seuils européens en deçà desquels l’étude environnementale et l’analyse coût bénéfice ne sont pas requises, les modalités de calcul des audits énergétiques, les systèmes de de management de l’énergie et l’obligation de rénovation énergétique. Il supprimerait même la mention des « secrets protégés par la loi » et la publication bisannuelle d’un rapport de financement relatif à ces nouvelles obligations européennes. Ce n’est pas admissible : il nous faut tirer parti de toutes les exemptions européennes existantes, afin d’éviter tout risque de surtransposition pour les entreprises et les collectivités. Je rappelle que le coût annuel de l’article 27 a été chiffré, dans l’étude d’impact du projet de loi Ddadue, à 5 milliards d’euros pour l’État

Le maintien d’une exemption pour les énergies d’appoint dans la transposition de la directive RED III de 2023 me paraît constituer une surtransposition. En effet, cette exemption permettrait l’attribution de certificats d’économie d’énergie à des dispositifs à des dispositifs utilisant des combustibles fossiles à titre d’appoint, ce qui va à l’encontre des objectifs de transition. Nous proposons donc de la supprimer pour aligner la transposition française sur les exigences européennes et envoyer un signal clair quant à la nécessité d’une sortie rapide des combustibles fossiles.

Je ne suis pas favorable à cette disposition, qui revient sur un aménagement du projet de loi Ddadue initial conforme à l’article 15 de la directive du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.

présenté par la Commission européenne le 26 février 2025. Nous proposons trois ajustements. Premièrement, limiter aux seules mesures dont le retour sur investissement est inférieur à trois ans, et non à cinq ans, les actions retenues dans le plan d’action issu de l’audit énergétique ou du système de management de l’énergie,

Cette harmonisation est d’autant plus nécessaire que les entreprises industrielles, notamment les électro intensives, sont déjà soumises à de nombreuses obligations en matière d’efficacité énergétique. De fait, elles doivent élaborer différents plans de performance énergétique pour bénéficier de taux réduits

la transposer ! L’abaissement des délais, pour ce qui concerne les investissements pris en compte dans le plan d’action, ou leur allongement, pour ce qui est de la transmission de ce plan à l’autorité administrative, introduirait de la complexité par rapport aux autres dispositions de l’article 27. Il nous faut conserver des délais uniformes

Afin d’assurer la pleine conformité de notre droit avec celui de l’Union européenne, il n’est pas exclu que des ajustements, à la fois limités et techniques, soient nécessaires. La majorité de ces éventuelles modifications pourrait se faire dans le cadre de cette habilitation. Par ailleurs, cette demande

il est toutefois nécessaire d’adapter cette exigence à certaines catégories de bâtiments : ceux qui sont situés dans un périmètre de protection patrimoniale et architecturale,

L’article 5 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments vise à imposer aux États membres de fixer des exigences minimales de performance énergétique.

Alors que ces sites souffrent déjà d’un déficit de compétitivité important, l’obligation qui leur est imposée de réaliser des économies d’énergie dans les bureaux et les entrepôts détourne des ressources humaines et financières de projets de décarbonation plus pertinents. Aussi, cet amendement a pour objet d’exempter certains bâtiments, notamment sur les sites industriels, des obligations minimales de performance énergétique imposées au travers de l’article L. 174 1 du code de la construction et de l’habitation.

retient déjà les exemptions européennes à l’obligation de rénovation énergétique des bâtiments publics prévue dans la directive du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique. D’autre part, l’article L. 174 1 du code de la construction et de l’habitation

de sa cohérence avec le droit européen, la fin de la vente des voitures neuves à moteur thermique en 2035. La suppression de cet article, si le Sénat

serait comprise comme un signal politique, en ce qu’elle n’aurait pas formellement d’incidence sur la réalité de la mesure, et comme un encouragement pour tous ceux qui se refusent à prendre au sérieux l’urgence climatique et l’indispensable arrêt, à terme, des carburants fossiles.

retarder encore notre mutation industrielle. Notre amendement vise donc à préserver la tenue de cette ambition européenne.

relatif aux émissions de CO2 par les constructeurs automobiles. Le fait est que cette modification législative n’emporte pas de conséquences juridiques dans la mesure où le règlement est d’application directe.

Il faut fournir cette flexibilité, sans quoi les constructeurs, qui ont consenti de lourds investissements dans l’électrification de leur gamme et qui sont néanmoins confrontés à une demande de véhicules électriques actuellement atone, se retrouveront dans une situation impossible. Nous assumons

explication de vote. Une fois n’est pas coutume, monsieur le ministre, nous partageons votre propos et nous vous remercions de cette clarification salutaire.

ou si les « spécificités du projet industriel de l’exploitant […] le justifient ». L’objectif de ces dispositions est de donner de la visibilité aux exploitants d’aéroport s’ils doivent mener des investissements qui ne seront amortis que sur une longue durée. C’est en particulier le cas à Nantes Atlantique : il est nécessaire que l’appel d’offres soit attractif si nous voulons éviter qu’il ne soit encore abandonné, faute de concurrence. nous avons veillé à ce que l’ART soit impliquée dans toutes les étapes du processus, que ce soit en cas de renouvellement de la concession ou de projet industriel spécifique justifiant un contrat de dix ans. Nous concilions ainsi vision stratégique et protection des usagers.

l’Autorité, en revanche, de veiller à ce que la durée du contrat et le niveau des redevances soient cohérents avec le projet. Cet amendement explicite opportunément le partage des tâches entre l’ART, d’une part, et l’État

le sénateur Vincent Capo Canellas le sait. Au sein même du présent article, de nombreux ajustements sont prévus. Je vous rappelle, par ailleurs, que le dispositif de régulation économique des aéroports a fait l’objet d’une réforme profonde en 2024.

: La parole est à M. le ministre. Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour l’État de solliciter plusieurs avis auprès de l’Autorité de régulation des transports. Les procédures de mise en concession des aéroports sont des procédures complexes, pour lesquelles l’État concédant doit pouvoir utiliser, y compris en cours d’instruction, toutes les possibilités offertes par le code de la commande publique. La rédaction issue des travaux de la commission permet à l’État de consulter

de régulation économique (CRE) du candidat retenu, plutôt que sur ceux de l’ensemble des candidats. En effet, l’ART n’a pas les moyens de rendre un avis circonstancié sur les avant projets de tous les candidats à une telle procédure. Notre commission a d’ailleurs dénoncé à de nombreuses reprises le niveau insuffisant de sa dotation budgétaire. Il ne serait donc pas souhaitable d’alourdir trop fortement son plan de charge dans ce contexte. De surcroît, l’ART est une autorité de régulation ; son rôle n’est pas celui d’une société de conseil ou d’ingénierie. en contrepartie, nous avons prévu que l’ART se prononce sur le cahier des charges de la concession : son intervention en amont des offres des candidats est opportune, puisque la réponse respective de chacun d’entre eux dépend largement de la façon dont ledit cahier des charges est conçu. Je suis donc défavorable à cet amendement qui vise à rouvrir à l’administration la possibilité de saisir pour avis l’ART sur l’avant projet de CRE de chaque candidat à un appel d’offres de concession aéroportuaire.

en particulier celles issues des systèmes embarqués dans les véhicules et celles provenant de prestataires de services comme Google Maps, Mappy, etc. – sont susceptibles d’être associées au conducteur et, dès lors, de […] constituer des données à caractère personnel selon la manière dont elles seront utilisées

Ce dispositif, qui a pour objet de mettre la France en conformité avec la révision en 2023 de la directive européenne relative aux systèmes de transport intelligents, dite directive STI, doit permettre d’améliorer la fluidité du trafic et de renforcer la sécurité routière. Si ce dispositif peut concerner des données à caractère personnel, il n’a pas pour finalité de permettre la collecte et le traitement de données associées à des personnes physiques identifiées de manière nominative.

de même nature que ceux qu’elle possède déjà en matière de données numériques multimodales, et notamment de données relatives aux transports collectifs. Bien que l’article 30 reprenne pour l’essentiel les pouvoirs dont dispose déjà l’ART concernant les données numériques multimodales pour les étendre au champ des données numériques routières, il ne prévoit pas de pouvoir de sanction. Il s’agit donc ici de préciser les obligations mises à la charge des détenteurs et utilisateurs de données, par référence aux dispositions des règlements délégués pertinents, et à octroyer à l’ART un pouvoir de sanction en cas de manquement. L’adoption de cet amendement permettrait, dans un souci de cohérence, d’aligner le régime des données numériques routières le régime applicable aux données numériques multimodales, et d’assurer l’effectivité du pouvoir de recherche et de constatation de manquements prévu aux alinéas 18 et 19 de l’article 30, pouvoir qui serait privé d’utilité réelle si l’ART ne pouvait sanctionner les manquements correspondants. Quel est l’avis de la commission ? Je ne suis l’avis de la commission ? Je ne suis pas favorable à cet amendement, et ce pour deux raisons. D’une part, le Conseil d’État a estimé, dans son avis sur le projet de loi, que les obligations mises à la charge des détenteurs

sans méconnaître le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. En pratique, il sera certainement nécessaire de repréciser les contours du dispositif d’ici à quelques années, à la lumière des premiers retours d’expérience, avant d’être en mesure de créer un pouvoir de sanction. D’autre part, les obligations de fourniture de données prévues par cet article reposent sur un champ d’application très large, pour ce qui est tant des données concernées que du périmètre des acteurs assujettis, lequel comprend notamment des gestionnaires routiers, donc en particulier des collectivités territoriales, des fournisseurs de services d’information sur les déplacements, ou encore des constructeurs automobiles. Or un certain nombre de ces acteurs, à commencer par les collectivités territoriales, évidemment, auront besoin de temps pour adapter leurs outils numériques et se mettre en conformité avec la directive. avec la directive. Pour toutes ces raisons, et afin de ne pas mettre davantage de pression sur les collectivités territoriales, je recommande d’attendre la maturité du dispositif et de l’écosystème avant de doter l’ART d’un pouvoir de sanction. Avis défavorable.

de la Cnil, qui m’a confirmé que le fait de la solliciter un avis conforme, c’est à dire un avis contraignant pour le pouvoir réglementaire, était contraire à sa doctrine d’intervention comme à la jurisprudence. Une telle mesure représenterait en outre une charge administrative supplémentaire pour ses services d’instruction, dans un contexte de moyens déjà contraints.

La réécriture de cet article conduit à confier au gestionnaire de l’infrastructure et aux exploitants ferroviaires la charge de définir les tâches critiques pour la sécurité et les fonctions liées à la sécurité, ainsi que de déterminer le personnel chargé d’exercer Ce rôle était jusqu’à présent dévolu à l’État, par voie réglementaire, et à l’Établissement public de sécurité ferroviaire, et non aux entreprises elles mêmes ; L’adoption de deux amendements du rapporteur a permis d’apporter quelques garanties en ce domaine, et nous nous en félicitons. Une telle modification des règles pose néanmoins un problème d’équité : un même métier pourrait faire l’objet de règles différentes, à défaut d’unification par le législateur. Voilà les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article.

les États membres n’ont plus la possibilité de définir ces tâches : il incombe à chaque entreprise ferroviaire d’identifier les tâches critiques pour la sécurité et les fonctions liées à la sécurité, déterminer le personnel chargé de les exercer. Cet amendement de suppression mettrait notre droit interne en contradiction avec le droit européen, lequel est de surcroît, en l’espèce, d’application directe. Cette suppression n’aboutirait donc qu’à affaiblir la clarté et la lisibilité du droit, au détriment des salariés du secteur J’ajoute que je partage les préoccupations de l’auteur de l’amendement : cette harmonisation des règles ne doit avoir aucun effet négatif ni sur la sécurité ferroviaire ni sur les droits des travailleurs. cependant que cette nouvelle approche de la définition des risques par les opérateurs ferroviaires devrait leur donner la possibilité de mieux s’approprier les règles de sécurité. De plus, l’Établissement public de sécurité ferroviaire m’a expressément indiqué être « vigilant quant à la manière [dont] les exploitants appliquent la nouvelle réglementation européenne

Il ne me semble en effet pas souhaitable que n’importe quel médecin ou psychologue, éventuellement peu au fait des spécificités du secteur ferroviaire, puisse se prononcer sur l’aptitude du personnel ferroviaire. De surcroît, les modalités d’évaluation de l’aptitude étant très strictement encadrées par le droit européen, il est logique que les professionnels de santé concernés aient été formés à la façon dont ils doivent mener l’examen en question pour se conformer à la réglementation.

Le risque inondation est en France le premier des risques naturels ; il va s’intensifiant avec le changement climatique. Les collectivités sont pleinement associées tout au long des travaux de révision de ces plans, comme le prévoit la loi. Cette association en continu est préférable à une consultation intervenant à la fin du processus sur la base d’un dossier déjà bouclé. Or l’ajout d’une consultation supplémentaire des collectivités après la consultation du public, par la commission, ne ferait qu’allonger le délai de révision sans réelle plus value, retardant d’autant la mise en œuvre des mesures de prévention. Au moment où nous cherchons collectivement à accélérer le déploiement des projets de prévention des inondations, cette nouvelle consultation irait à l’encontre d’un tel objectif que je sais – ou

il ne me semble pas souhaitable de supprimer une telle étape de consultation. Les élus locaux sont en première ligne en matière de gestion des inondations, comme l’actualité ne cesse de le démontrer, et les PGRI ont des incidences réelles sur les documents d’urbanisme. Une association en continu des collectivités territoriales au cours du processus d’élaboration du PGRI est bien entendu souhaitable, comme vous l’avez souligné, mais cela n’exclut pas, à mon sens, que leur soit soumise la version finale du projet de PGRI, intégrant notamment les modifications apportées à la suite de la consultation du public.

Depuis près d’un an, nous avons donc été plusieurs à être sollicités, dans nos territoires, et à nous mobiliser pour que la France aligne son calendrier sur celui de l’Union En septembre 2024, le Gouvernement a publié un avis afin d’acter l’inapplicabilité de l’interdiction prévue à compter de 2025 ; un premier pas Mais le droit français reste en contradiction avec le règlement européen. Il s’agit donc, par cet article, de mettre fin à cette incohérence afin de garantir l’harmonisation juridique qui est l’objet même de ce projet de loi.

Cette avancée est importante pour rassurer les industriels et leurs clients et leur permettre d’envisager les prochaines années avec davantage de sérénité. Permettez moi enfin d’anticiper sur la discussion de l’amendement à venir en vous invitant, mes chers collègues, à maintenir cet article 39 .

une disposition qui date des années 1950. Or cette restriction entre en contradiction avec deux principes fondamentaux de l’Union européenne : la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement. La Commission européenne a donc adressé une lettre de mise en demeure à la France

plus grande mobilité professionnelle, y compris entre la France et des pays situés hors de l’Union européenne. Sans doute le président Mouiller sait il déjà tout cela et soutiendra t il cet amendement du Gouvernement

Le présent amendement de coordination juridique vise à apporter deux modifications aux dispositions prévues à l’article 41. D’une part, il tend à déplacer les dispositions relatives aux pouvoirs de police sanitaire de l’Agence nationale nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en matière de dispositifs médicaux (ANSM) au début du chapitre du code de la santé publique relatif à la lutte contre les ruptures d’approvisionnement de dispositifs médicaux. D’autre part, il vise à créer dans le code de la santé publique un nouveau chapitre relatif à la lutte contre les ruptures d’approvisionnement de dispositifs médicaux de diagnostic et à y déplacer les dispositions de l’article 41 relatives aux pouvoirs de police sanitaire de l’ANSM dans ce secteur.

On ne peut pas dire que j’aie été entendu, si l’on en juge par le mauvais signal envoyé à l’électromobilité, les reculades pour la mise en œuvre de la régulation de la durabilité des entreprises, le bridage du développement des énergies renouvelables ou encore le déséquilibre opéré au détriment de la biodiversité. Le groupe écologiste désapprouve fortement cet « apport » sénatorial,

nous sommes de ceux qui estiment que l’Europe est aussi facteur de progrès et que nous en sommes toutes et tous comptables. La législation européenne, que ce soit au travers de règlements

modifié, l’ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. La parole

aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, présentée